Monsieur le ministre,

sanitaire a autorisé le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, le CPSTI, ainsi que les instances de gouvernance des régimes de retraite complémentaires, des professionnels libéraux et des avocats à mobiliser une fraction de leurs réserves financières pour financer des aides exceptionnelles destinées aux cotisants de ces régimes. À l'instar des dispositifs d'exonération applicables aux aides versées par le Fonds de solidarité institué par l'ordonnance du 25 mars 2020, l'article 3 du présent projet de loi de finances prévoit que les aides ainsi versées par le CPSTI sont exonérées de tout impôt sur les bénéfices et des cotisations sociales associées. Le même article prévoit par ailleurs que les effets du versement de ces aides pour la détermination du régime d'imposition applicable au bénéficiaire sont neutralisés. Le présent amendement vise donc à appliquer ce dispositif d'exonération à l'ensemble des aides versées par les sections professionnelles de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et par la caisse nationale des barreaux français, en application de l'article 10 de la loi du 17 juin 2020 précitée.

Cet article 3 vise à créer un crédit d'impôt dans le cadre du plan de relance en faveur de la rénovation énergétique. Ce programme de rénovation énergétique

On ne peut que regretter que l'acquisition et la pose de chaudières gaz à très haute performance énergétique ne figurent pas parmi la liste des travaux éligibles à cette nouvelle aide.

revanche, pour répondre à la question de M. Capus, les entreprises qui réalisent elles-mêmes les travaux sur leurs bâtiments sont en effet éligibles au crédit d'impôt, à condition de pouvoir démontrer les coûts liés à l'achat et à la pose des fournitures.

c'est la réduction des consommations d'énergie ; la cible, ce sont les PME et TPE ; la technique, ce sont les chauffe-eau thermodynamiques et les pompes à chaleur ; les moyens, c'est l'extension de MaPrimeRénov'.

fixes de classe énergétique supérieure ou égale à A+ pour la performance de chauffage, avec quelques précisions concernant les économies d'énergie qui peuvent résulter de l'utilisation de cet appareil.

à M. Pierre Cuypers. Dans l'hypothèse où les chaudières à très haute performance énergétique ne seraient pas intégrées au crédit d'impôt sur la rénovation énergétique des bâtiments tertiaires, le présent amendement a pour objet de reprendre la terminologie exacte de ce type d'équipements, prévue pour le crédit d'impôt pour la transition énergétique. M. Pierre Cuypers. Il s'agit toujours de conforter le crédit d'impôt en l'étendant aux dépenses relatives à l'acquisition et à la pose de chaudières à très haute performance énergétique hors fioul.

? Ces amendements identiques visent à apporter un soutien public au développement de l'électromobilité en entreprise, en rendant éligibles au crédit d'impôt des dépenses

effet, les crédits prévus à hauteur de 95 millions d'euros sur deux ans dans le plan de relance visent notamment à financer des diagnostics et un accompagnement à la transition écologique, pour les professionnels, artisans, commerçants et indépendants. La commission demande donc le retrait

Guillaume Gontard. Cet amendement vise à faciliter la prise de congés des agriculteurs, en augmentant le montant du crédit d'impôt permettant de financer le recours au service de remplacement. Actuellement, ce crédit d'impôt permet aux éleveurs et aux paysans contraints à une présence quotidienne dans leur ferme de bénéficier d'un financement égal à 50 % des dépenses de remplacement pour congé,

Mme Sylvie Vermeillet. L'article 3 du PLF prévoit des modalités déclaratives dérogatoires des sommes soumises au versement libératoire de l'impôt sur le revenu pour les micro-entrepreneurs bénéficiant du dispositif d'exonération de cotisations sociales mis en place par la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 2020 de finances rectificative pour 2020. Le présent amendement étend ces modalités déclaratives dérogatoires aux micro-entrepreneurs bénéficiant du dispositif d'exonération de cotisations sociales complémentaire introduit par l'article 6 du du PLFSS pour 2021, destiné à soutenir les entreprises affectées par les nouvelles mesures sanitaires prises pour faire face au rebond de l'épidémie, notamment par la mise en place d'un couvre-feu dans les zones d'alerte maximale, suivie d'un confinement sur l'ensemble du territoire. Quel

met à jour un certain nombre de méthodes d'évaluation de la valeur locative des établissements industriels et modifie le coefficient de revalorisation de la valeur locative de ces établissements. Voilà qui me donne l'occasion

milliard d'euros. Le groupe socialiste du Sénat tient à vous alerter, monsieur le ministre : la compensation pour les collectivités ne sera pas intégrale. Elle intègre, certes, la dynamique des bases, y compris en cas d'installation de nouvelles entreprises, mais elle sera calculée sur les taux de 2020, qui, cette année, sont gelés, comme les taux de la taxe d'habitation été en 2017. De plus, cet article pose, de manière plus générale, une question relative à la répartition de la charge fiscale en France entre les entreprises et les particuliers. Le Gouvernement continue de centrer l'imposition sur les ménages,

à 10 milliards d'euros. Cette baisse très importante, aux résultats incertains, n'est pas sans conséquence pour les collectivités locales, pour l'emploi et pour l'environnement, car, ici non plus, vous n'avez pas intégré de conditionnalité. En diminuant les impôts de production de l'ordre de 10 milliards monsieur le ministre, vous faites le choix d'une relance par l'offre, dans un contexte d'augmentation du chômage. Vous privilégiez, une nouvelle fois, cette politique, à l'efficacité contestable quand elle est conduite seule. Le plan de relance est déséquilibré, cet article en est la preuve. Le Gouvernement s'entête donc malheureusement dans une logique libérale,

prévoit la révision de l'évaluation de la valeur locative des établissements industriels et la modification du coefficient de revalorisation de la valeur locative de ces établissements, deux paramètres- les élus locaux le savent bien -qui n'ont pas été actualisés depuis leur détermination, en 1973, et qui ne sont plus adaptés à la réalité économique actuelle. Cette mesure pérenne permettra une réduction de moitié de la valeur locative de ces établissements, se traduisant également par une réduction de moitié des cotisations d'impôts fonciers pour environ 32 000 entreprises exploitant 86 000 établissements, et par un allègement des contributions dues par les entreprises au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties, la TFPB, et de la cotisation foncière des entreprises, la CFE. Cette mesure

remettant ainsi en cause 1,75 milliard d'euros de taxe foncière et 1,56 milliard d'euros de CFE. Si nous ne pouvons critiquer l'objectif de relance de la compétitivité des entreprises industrielles, alors que leur activité a été lourdement affectée par la crise sanitaire et que les impôts de production sont sept fois plus élevés en France qu'en Allemagne- et en moyenne deux fois plus que dans les pays de la zone euro -, cette baisse des impôts de production ne s'accompagne d'aucune baisse de la fiscalité nationale, en particulier de la contribution sociale de solidarité des sociétés, la C3S, pourtant jugée comme la plus nocive pour la compétitivité des entreprises par le Conseil d'analyse économique, le CAE. Cette baisse, qui s'inscrit dans une politique nationale de relance de l'industrie, doit être intégralement assumée par l'État, et non par les collectivités. Les pertes de recettes pour les communes et les EPCI seront compensées par un prélèvement sur recettes de l'État. La perte à compenser chaque année sera calculée sur la base des taux de CFE TFPB figés à leur valeur de 2020. En outre, le PLF pour 2021 prévoit de modifier les modalités de revalorisation des valeurs locatives des locaux industriels basée sur l'évolution de l'indice des prix à la consommation relatives aux locaux professionnels. Ainsi, contrairement aux annonces du Gouvernement, la compensation des pertes de ressources sur la base des taux figés et des bases quasi gelées remet en cause fortement le dynamisme des taxes foncières à la charge des établissements industriels. Par ailleurs, en continuant à remettre en cause la CFE et la taxe foncière après la suppression de la taxe d'habitation, l'État va aggraver l'affaiblissement financier et fiscal du bloc communal. Cette réduction des moyens financiers des communes et des intercommunalités fait peser un risque sur la reprise économique, en limitant la participation du bloc communal au plan de relance, alors que les communes et leurs EPCI plus de 65 % de l'investissement public local. En outre, l'idée selon laquelle la crise de l'industrie résulterait du niveau des impôts locaux est fausse : l'écart de compétitivité de l'ensemble des entreprises avec les autres pays européens provient surtout du poids des charges sociales, à près de 16 points de PIB. Le présent amendement vise donc à annuler la remise en cause de la CFE et de la taxe foncière perçues par le bloc communal à hauteur de 3,4 milliards d'euros. La

à aider les petites entreprises, ni le secteur de l'hôtellerie ni celui de la restauration. Les grands gagnants sont les grandes entreprises de l'énergie et de l'industrie, mais aussi les sociétés à forte intensité capitalistique, sans condition. Il en va comme pour la suppression de la taxe d'habitation d'habitation : le Gouvernement a voulu nous faire croire qu'elle bénéficierait aux ménages les plus modestes, alors que le bénéfice était beaucoup plus important pour les personnes les plus aisées. Cet article 4 est tout à fait dommageable. Les pertes pour les communes et les EPCI sont certes compensées par un prélèvement sur recettes de l'État, qui évoluera en fonction des bases, mais non en fonction des taux votés par les élus,

les industries de production et de distribution de fluides et d'énergie, pour 500 millions d'euros, et les entreprises d'entreposage et de transport, pour 300 millions d'euros.

préserver leurs ressources. Le présent article, en effet, instaure un prélèvement sur recettes de l'État. Cette modalité de compensation appelle deux observations. Premièrement, il eût été préférable et souhaitable de pouvoir bénéficier d'un dégrèvement, qui garantirait à l'euro près la compensation. Mais une telle mesure ne pouvait être envisagée, car elle aurait certainement constitué, au regard du droit européen, une aide de l'État. Deuxièmement, les conditions de calcul et d'évolution du montant des attributions qui sont versées au titre du prélèvement sur recettes préservent dans leur ensemble l'intérêt financier des collectivités locales.

Je plaide effectivement depuis longtemps, dans cet hémicycle, pour que les exonérations de taxe foncière sur le logement social et le logement intermédiaire soient véritablement compensées aux collectivités, ce qui n'est pas le cas. Pour le coup,

pas de combat. Nous sommes évidemment tous favorables au maintien de l'autonomie fiscale des collectivités territoriales. Nous sommes tous convaincus qu'il faut que les collectivités territoriales préservent leurs ressources. Toutefois, nous ne pouvons

Mme Gatel souligne également qu'il était possible d'envisager d'autres réformes, comme la suppression de la contribution sociale de solidarité des sociétés, la C3S. L'amendement qui vise à annuler la remise en cause de la CFE et de la taxe foncière perçue par le bloc communal à hauteur de 3,4

Je n'appuie pas toujours le Gouvernement- il m'arrive même parfois de le critiquer -, mais je suivrai M. le rapporteur général, qui a une position équilibrée.

L'enjeu est non pas de remettre en question une mise à jour nécessaire de ces paramètres qui datent de 1973, mais d'éviter une évolution trop brusque qui diminuerait de moitié les recettes fiscales qui y sont liées. Plutôt que d'imposer une réduction de moitié des taux d'intérêt actuellement en place, il conviendrait d'arriver à ces taux d'intérêt non pas pour 2021, mais pour 2022. 2022. Fonctionner par phase, avec une première diminution de 25 %, permettrait aux communes de ne pas ressentir trop brutalement cette réduction drastique. Certes, l'article prévoit également un prélèvement sur les recettes de l'État destiné à compenser pour les communes, les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre et la métropole de Lyon la perte de recettes résultant de la révision des taux d'intérêt. Le sens de cet amendement est double : il permet à la fois une réduction progressive sur deux années des taux d'intérêt pris comme base de calcul pour la taxe foncière sur les propriétés bâties et pour la cotisation foncière des entreprises, tout en maintenant le principe de la réduction des charges fiscales pour les entreprises. La réduction progressive des taux d'intérêt se ferait en deux étapes. Pour l'année 2021, ce taux d'intérêt serait de 6 pour les sols et terrains, contre 8 % actuellement, et de 9 % pour les constructions et installations, contre 12 % actuellement, soit une diminution de l'ordre de 25 %. Pour l'année 2022, les taux d'intérêt atteindraient la valeur souhaitée par l'administration, à savoir 4 % pour les sols et terrains et 6 % pour les constructions et installations, soit une nouvelle réduction de 25 % par rapport aux taux appliqués que l'on peut retrouver à l'article 310 L de l'annexe 2 du code général des impôts. La compensation prévue par l'État s'adapterait également, n'étant pas immédiatement de moitié, mais d'abord d'un quart pour 2021, puis de la moitié pour 2022. Il ne faut pas que, à terme, les ressources fiscales des collectivités s'en trouvent diminuées, sans quoi leur capacité d'investissement serait durablement ce qui est d'autant plus important pour les communes touristiques, telles que les communes supports de station de montagne. Cette compensation se doit d'être durable dans le temps. Les communes sont plus que jamais confrontées à des tensions financières avec une diminution croissante de leurs recettes, alors que leurs missions sont toujours aussi nombreuses. Les communes touristiques assument d'ailleurs des charges plus lourdes du fait de l'investissement nécessaire à l'attractivité touristique, faisant de la compensation un levier indispensable. Le contexte sanitaire a rendu l'économie fragile, mais également les collectivités, qui sont directement affectées. Les communes touristiques le sont d'autant plus qu'elles sont soumises à des dépenses plus importantes.

plus important à mes yeux, il vise à corriger à la marge le dispositif de compensation de la taxe d'habitation votée l'année dernière. Il existe en effet des effets de bord sur les taxes additionnelles, notamment pour les établissements publics fonciers et les syndicats non fiscalisés.

En l'état, la réduction de la CFE et de la TFPB des entreprises industrielles est compensée par un prélèvement sur recettes qui prend en compte l'évolution des bases imposables, mais les taux sont gelés

? Cet amendement a pour objet que la perte de base prise en compte pour le calcul de la dotation de compensation instituée par l'article 4 au profit des collectivités du bloc communal soit calculée avant la mise en oeuvre de l'abattement prévu à l'article 1472 A du code général des impôts. du Gouvernement ? Cet amendement est satisfait : je confirme que l'abattement de 25 % s'appliquant conformément à la loi à la base d'imposition n'est pas pris en compte pour calculer la perte de base d'imposition servant au calcul de la compensation prévue à l'article 4. Le dispositif de compensation proposé sera même favorable aux collectivités de Corse, puisqu'il aboutira à rafraîchir le taux de compensation, en compensant sur la base du taux de 2020 une partie des bases qui était jusqu'alors compensée avec le taux historique de 1994.

Cet amendement vise donc à conditionner la baisse de CFE et de taxe foncière à des obligations en matière sociale, environnementale et fiscale, pour les entreprises dont la taille correspond ou excède le seuil européen de l'entreprise moyenne. Il a pour objet la mise en place de plusieurs obligations conditionnant l'éligibilité à la baisse d'impôt : non-versement de dividendes ; non-détention d'actifs dans un paradis fiscal ; remise d'un rapport annuel faisant état de la trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l'horizon de 2030, pour atteindre les objectifs fixés par le plafond national des émissions de gaz à effet de serre ; enfin, mise en place d'un plan de vigilance. Le non-respect d'au moins une de ces quatre obligations entraînerait un remboursement du bénéfice de la baisse de CFE ou de taxe foncière et au paiement d'une amende pouvant atteindre 5 % du chiffre d'affaires mondial consolidé de la société. ? Le dispositif de l'article 4 ne permet pas d'introduire ce type de contrepartie. En effet, il ne prévoit pas en tant que telle une une baisse d'impôts : il fixe une nouvelle modalité de calcul de la valeur locative d'un local industriel. Or cette valeur locative est attachée à un local, elle est donc indépendante de l'entreprise

Cet amendement a pour objet de majorer de manière temporaire les coefficients d'amortissement dégressif. Il vise donc à encourager l'investissement des entreprises,

vous le savez, j'ai eu l'occasion de dire combien, dans la période de relance, il est important de définir et de choisir des mesures temporaires d'accélération et de dynamisation de notre économie. Certes, des entreprises

Si une entreprise ne déduit pas son amortissement une année, elle en perd le bénéfice les années suivantes. Celles qui ont eu une forte perte de chiffre d'affaires à la suite de l'arrêt d'activité ont eu un bénéfice d'exploitation réduit et la déduction de l'amortissement créera un déficit.

PME aux investissements des entreprises industrielles et tertiaires réalisés en matière d'efficacité énergétique, dès lors que les économies générées sont suffisamment significatives et garanties, ainsi qu'en matière de chaleur renouvelable ou de récupération. Le dispositif serait par ailleurs étendu jusqu'au 31 décembre 2023.

bénéficient d'un dispositif de suramortissement pour certains biens acquis à l'état neuf, mécanisme qui leur permet une déduction accélérée de la valeur de ces biens inscrits à l'actif immobilisé. Ce dispositif qui vise à inciter les entreprises à s'équiper en biens stratégiques exclut expressément les biens reconditionnés et défavorise les PME qui s'engagent dans une démarche d'achat de biens reconditionnés. Si le plan de relance prévoit bien un soutien à l'informatisation des entreprises et une enveloppe en faveur de l'économie circulaire et du réemploi, nous n'avons pas, à ce stade, le détail de ce qui sera réellement éligible. Notre amendement vise donc à étendre le dispositif de suramortissement existant aux équipements reconditionnés. Cette mesure permettra aux TPE-PME bénéficiaires de s'équiper en biens informatiques, notamment le petit matériel mis à la disposition des salariés pour favoriser le travail à distance- ordinateur, clavier, etc. moins chers, et avec une empreinte environnementale plus faible, en favorisant la création d'emplois en France, les reconditionneurs étant majoritairement des TPE-PME françaises. C'est vraiment

tend plus spécifiquement à élargir le bénéfice de ce mécanisme, qui a été introduit dans la loi de finances pour 2019, au secteur agricole. L'objectif, qui est, je pense, largement partagé ici, est d'accélérer la modernisation de nos exploitations agricoles. Nous le savons tous, les agriculteurs investissent de plus en plus dans les nouvelles technologies, notamment la robotique et l'intelligence artificielle. Il convient de les encourager à accélérer en la matière. La parole est à M.

pour l'acquisition et l'installation d'infrastructures de recharge des véhicules terrestres en carburant alternatif ouvertes au public. Je rappelle qu'un amendement similaire avait été adopté au Sénat dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances rectificative de juillet 2020, avec, je le rappelle également, l'avis favorable du Gouvernement. cet amendement est similaire à celui proposé par le Gouvernement pour l'avitaillement des navires, dans le cadre de la loi de finances initiale pour 2019.

au cours de l'été dernier dans le cadre du troisième projet de loi de finances rectificative, ici au Sénat. L'article 39 C du code général des impôts instaure un mécanisme de suramortissement fiscal pour certains investissements réalisés par les armateurs, afin d'inciter les compagnies maritimes à acquérir des navires utilisant des sources d'énergie plus respectueuses de l'environnement. Or vous proposez, avec cet amendement, de mettre en place une déduction fiscale pour l'acquisition et l'installation d'infrastructures de recharge des véhicules terrestres en carburant alternatif ouvertes au public. Autant sur la question

l'étendue du dispositif que vous proposez présente un risque de non-conformité avec la réglementation européenne des aides d'État. Par ailleurs, nous préférons, pour ce qui concerne le développement de ces infrastructures, intervenir directement par des crédits, plutôt que par la politique fiscale.

avons un objectif dans ce pays, à savoir déployer pour 2021 plus de 100 000 bornes d'électricité. Si l'on ne se prend pas par la main, on n'y arrivera jamais ! Je mets

je serais intéressé par entendre la commission et le Gouvernement, pour savoir celui qui, sur le fond et sur la forme, est le plus adéquat, mais, dans tous les cas, c'est le même objectif : mettre un terme à cette inégalité.

de fonctionnement de structures d'accueil d'enfants, ainsi que des dépenses de services à la personne. Il s'agit en fait d'inciter les entreprises à aider leurs salariés, en complément des dispositifs fiscaux dont ces derniers peuvent déjà bénéficier à titre individuel. C'est une manière,

du Gouvernement ? C'est un sujet complexe que celui de l'accès ou non des indépendants au crédit d'impôt famille. Je tiens à rappeler que l'équilibre financier des entreprises de crèche repose sur trois piliers une part payée par les familles ; une part payée par la branche famille et une part payée par des tiers financeurs, c'est-à-dire des entreprises qui réservent des places pour leurs salariés et bénéficient à ce titre du Cifam, ou des collectivités qui versent des subventions. La proposition qui est portée par tous ces amendements, quel que soit leur périmètre, ne nous paraît en réalité pas avantageuse pour les indépendants, puisque, pour bénéficier du Cifam, ceux-ci devraient acquitter la part de tiers financeur des crèches.

Par ailleurs, il faut préciser que le Cifam soutient les entreprises qui proposent une offre de garde à leurs salariés en vue de l'amélioration de leurs conditions de vie. Ce dispositif a été adopté en PLF pour 2004 pour inciter les entreprises à prendre des mesures en faveur de leurs salariés ayant des charges de famille et des enfants en bas âge. Or la proposition que vous portez, si elle était adoptée, conduirait notamment à financer l'action sociale pour soi-même au travers d'un dispositif fiscal dédié aux entreprises créant de l'emploi salarié, ce qui n'est pas l'objectif, ou en tout cas pas l'esprit du dispositif du Cifam. Il existe une différence entre un employeur qui met en place une politique sociale d'accueil des jeunes enfants pour ses salariés et un indépendant qui réserverait et financerait lui-même sa place de crèche d'entreprise uniquement pour son propre enfant, c'est-à-dire, si je puis dire, à son seul bénéfice. il est admis par la doctrine administrative que le fait pour les crèches ou les haltes-garderies d'accueillir également les enfants du personnel non salarié d'une même entreprise, comme les gérants non-salariés ou les professions libérales, ne remet pas en cause le bénéfice du crédit d'impôt, ce qui répond, je crois, à une partie au moins de vos préoccupations. Enfin, j'ajoute que les membres des professions libérales et les artisans bénéficient déjà d'un crédit d'impôt pour dépenses de garde d'enfants de moins de 6 ans, prévu à l'article 200 B du code général des impôts.

le fait générateur de la politique familiale, c'était l'enfant, non le statut des parents. Or, dans votre réponse, il y a une totale confusion entre les deux. D'ailleurs, il est assez révélateur que vous n'ayez pas employé une seule fois le mot « famille » ; vous vous référez plutôt à la politique sociale ... Par conséquent, je voterai ces amendements, car je ne vois pas pourquoi il y aurait une inégalité de traitement des enfants en fonction de la profession des parents.

On sait que ces derniers ont été bénéficiaires, bien malgré eux, d'ailleurs, de la chute significative du nombre de sinistres couverts, en particulier en assurance dommages et santé-prévoyance. L'idée est que le produit de cette taxe soit mis à profit pour soutenir les actions en faveur des petits commerces, TPE et PME.

à 9 milliards d'euros. Bpifrance a confirmé cette estimation, en évaluant, de son côté, la perte d'exploitation consolidée du secteur des cafés, hôtels, restaurants et discothèques entre 7,3 milliards et 9,3 milliards d'euros, en fonction des différentes hypothèses de reprise. Si certains accords ont pu être trouvés entre restaurateurs et assureurs, les professionnels de l'assurance sont encore trop nombreux à opposer des refus catégoriques aux demandes de prise en charge des pertes d'exploitation pour une fermeture administrative, alors même que des polices d'assurance le prévoient expressément. Cette situation de blocage conduit à une multiplication des contentieux, dont l'issue sera probablement tardive. La question de la prise en charge des pertes d'exploitation est pourtant essentielle pour la survie de ces entreprises. L'urgence de la situation appelle une réponse immédiate de la part des assureurs, qui doivent intervenir de manière plus ambitieuse au nom de la solidarité nationale. Le produit de cette taxe devrait être mis à profit pour soutenir les actions en faveur des professionnels du secteur, qui se trouvent aujourd'hui dans une situation économique sans précédent.

C'est un engagement que le Sénat a pris très tôt, dès le début de la pandémie, avec un large consensus. Nous n'avons pas attendu, puisque, début juin, ici même, une proposition de loi a été adoptée à l'unanimité des suffrages exprimés pour appeler à la mobilisation des assureurs, afin de faire face aux garanties, notamment pour couvrir les charges fixes des entreprises dans ces conditions. La participation des assureurs se justifie pleinement.

Le Parlement a demandé au Gouvernement, qui a donné suite, un rapport sur l'évolution de la sinistralité. Ce rapport précise qu'un effet se dégage en avril et en mai, puisque l'on constate une baisse des sinistres de 25 %, toutes catégories confondues, sauf pour l'assurance non-vie.

a pu y avoir un effet de report à ne pas négliger. Ils se sont engagés sur une contribution au financement de l'économie, mais je pense que, dans les circonstances que nous avons connues, et que nous connaissons encore, une contribution exceptionnelle peut-être sollicitée. En revanche, je ne crois pas que toucher aux réserves de capitalisation soit une bonne idée, parce que cela remettrait en cause à la fois la prévisibilité et les normes auxquelles les compagnies d'assurances doivent obéir. En outre, ces réserves de capitalisation constituent, pour une part, la partie privée

le Gouvernement n'a pas considéré comme opportun ni même justifié de procéder à un prélèvement particulier sur les assurances. Sur la méthode, j'ai eu l'occasion de dire que les modalités de prélèvement proposées par ces quatre premiers amendements nous paraissaient contrevenir, ou du moins ou du moins présenter des difficultés par rapport aux règles prudentielles. Sur le fond, nous avons la volonté de continuer à travailler avec le secteur, ce qui m'amènera à m'opposer aussi tout à l'heure à l'amendement présenté par M. le rapporteur général. Mais, dans l'attente, sur ces quatre amendements, je le répète, le

je propose que le Gouvernement se saisisse du travail qui a été réalisé ici. Il n'est certainement pas parfait, mais c'est une excellente base, parce qu'il s'intéresse uniquement aux crises pandémiques et au rôle

Monsieur le ministre, je suis sensible à vos arguments et je souscris aux éléments chiffrés que vous nous avez donnés. La Fédération française de l'assurance, que nous avons auditionnée, nous a également donné des arguments. Il n'empêche que nous souhaitons voir mise en place cette contribution exceptionnelle, au titre de la seule année 2020, à hauteur de 1 % du chiffre d'affaires sur les assurances dommages, ce qui doit produire de l'ordre de 600 millions d'euros. Quand Quand vous ajoutez ce montant aux contributions multiples et diverses du fonds de solidarité et à un certain nombre d'actions ou d'investissements au service de l'économie, et aux gestes extracontractuels faits par un certain nombre de compagnies, je pense que nous sommes sur la voie de la raison, tandis qu'un message fort

faut raison garder. Je ne suis pas un justicier ; j'essaie simplement de proposer, en responsabilité, l'approche la plus équilibrée possible. Je rappelle que les compagnies d'assurance vivent des primes et des cotisations que les Français paient.

Monsieur le ministre, que les contributions évoquées ne purgent évidemment pas le débat autour de la prise en charge des pertes d'exploitation et de la nature des contrats et des polices qui unissent les assureurs et leurs assurés. Je voulais l'ajouter, puisque j'avais eu l'occasion de le dire aussi

particulière d'entreprises que sont les assurances. On parle de « gestes », d'« abondements », et on les remercie presque pour cela ... Il me semble que les autres Français paient des impôts. Il appartient à à l'État, au Gouvernement et aux assemblées de décider quelle est la taxation, juste et légitime, qui doit être appliquée aux assurances dans le contexte particulier de cette crise. Je le répète, je suis très surpris. On a l'impression que l'on traite de relations contractuelles,

M. Philippe Dominati, pour explication de vote. Je voudrais faire une remarque et obtenir une précision. Monsieur le rapporteur général, je suis particulièrement hostile à toute taxation nouvelle, surtout lorsqu'elle est exceptionnelle, parce que rien ne garantit qu'elle le reste

répercutée sur les usagers et sur les clients des assurances. Pour ma part, j'aimerais avoir la certitude qu'il n'y aura pas automatiquement un tel report, d'autant que, le Gouvernement n'étant pas favorable à cette solution, il n'y aura pas de contrôle de la part de l'exécutif vis-à-vis

le résultat du scrutin. Voici, compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence,

de 30 % à l'impôt sur les sociétés pour les investissements dans des diagnostics d'audit de cybersécurité ou l'acquisition de solutions de protection des données ou du système informatique des entreprises.

créer, en faveur des commerces de proximité, une contribution exceptionnelle de la part des grandes et moyennes surfaces, ainsi que des plateformes de commerce électronique.

à titre exceptionnel et pour la seule année 2020, de taxer le chiffre d'affaires réalisé par les grandes entreprises de vente de biens ou de fourniture de services

financier d'amortissement utile pour les entreprises. L'amendement vise à augmenter la durée

aurait un coût pour les finances publiques extrêmement important, et que, par ailleurs, la proposition, telle qu'elle est rédigée, nécessiterait de « tunneliser »- pardonnez ce barbarisme -les déficits des entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés, afin d'identifier ceux afférents à la gestion d'un patrimoine mobilier ou immobilier, accroissant ainsi la complexité du dispositif.

Il y a deux problèmes. Le premier tient à la difficulté de distinguer, au sein des entrepôts, les biens qui sont destinés à la vente en ligne et ceux qui sont destinés à la vente physique. Le second concerne le risque de réorganisation sur les chaînes d'approvisionnement, car, pour les acteurs du commerce en ligne qui sont visés,

J'ai conscience qu'il existe un problème sur le niveau et surtout l'équilibre d'imposition entre les opérateurs. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle

pour la cinquième année consécutive, avec le même amendement, que le Sénat a systématiquement adopté, à la quasi-unanimité ! Il s'agit de faire en sorte que les exonérations de taxe sur le foncier bâti accordées aux bailleurs sociaux

C'est d'autant plus urgent, mes chers collègues, que l'année prochaine, la taxe d'habitation disparaîtra et qu'une grande bascule s'opérera : il ne restera plus que le foncier bâti pour les communes.

À ce stade, l'avis du Gouvernement est toujours défavorable sur l'amendement que vous avez déposé, pour des raisons essentiellement budgétaires, même si, vous le savez, la question de la compensation ou de la non-compensation

S'agissant de la réforme de la taxe d'habitation, il suffit de regarder le montant des douzièmes perçus par les collectivités au cours de l'année actuelle, alors que 80 % des ménages ne payent plus cette taxe : vous constaterez ainsi aisément que la compensation ou les dégrèvements dont bénéficiaient un certain nombre de contribuables qui ne payaient pas la taxe d'habitation pour des raisons liées à la faiblesse de leurs revenus ont été intégrés dans le modèle de compensation.

notamment des contraintes européennes. Je tiens cependant à vous rassurer, mon cher collègue : dans le cadre de la commission mixte paritaire conclusive

titre, observer un ralentissement du commerce physique. Or la taxe sur les services numériques concerne, non pas directement cette assiette, mais bien les seuls revenus tirés de l'intermédiation et de la vente de données à des fins publicitaires.

France », égal à 10 % des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement affectés à la réalisation de produits fabriqués

globale. Votre dispositif constitue une sorte de crédit d'impôt sur les salaires versés, avec une condition supplémentaire sur l'origine de la valeur ajoutée des produits.

C'est la raison pour laquelle l'amendement vise à modifier le code général des impôts, afin de prévoir ce cas très particulier de restructurations « intercalaires » intervenant avant la deuxième fusion.

comportementale. Une taxe écoresponsable s'appliquerait pour les consommateurs du e-commerce, en fonction de la valeur du colis. Ce dispositif incitatif prévoit que les transactions donnant lieu à la livraison physique de biens en un lieu autre qu'un point de retrait ou un magasin soient assujetties à une écocontribution écocontribution forfaitaire en fonction d'un barème lié au montant de la commande. L'objectif est de rétablir la justice.

Avec cet amendement de suppression, nous profitons de la volonté du Gouvernement de défiscaliser les réévaluations libres d'actifs pour évoquer le sujet important de la compatibilité écologique.

Concrètement, il faudrait intégrer dans leur comptabilité les impacts de l'activité économique sur l'environnement et le monde social. Il faut compter différemment ce qu'est une création de valeur, laquelle ne peut plus se réduire à de la valeur financière. l'article 5 prévoit de neutraliser la position sur la réévaluation libre des actifs, mécanisme qui s'inscrit dans une vision purement actionnariale : quand on réévalue des actifs au prix du marché, on compte du point de vue de l'actionnaire qui veut évaluer sa richesse au moment , , non du point de vue de l'entreprise, qui comptabiliserait le montant d'intrant initial pour son activité productive. Il faut donc une autre comptabilité, réformée. C'est pourquoi nous refusons cette mesure non conditionnée, qui consiste à créer de la valeur selon une logique actionnariale.

l'article 5, lequel vise à permettre une neutralisation temporaire des conséquences fiscales d'une réévaluation, pour permettre aux entreprises d'améliorer leur bilan et de renforcer, ainsi, leur capacité de financement. Il ne s'agit donc pas d'une exonération de la plus-value. Celle-ci est bien réintégrée, mais elle l'est selon des modalités différenciées, selon qu'il s'agit d'un actif amortissable ou non.

Afin de préparer la reprise, il est indispensable de venir consolider les fonds propres des entreprises. Le projet de loi de finances pour 2021 prévoit la réévaluation des actifs corporels et financiers, ainsi que l'exonération de la plus-value réalisée par les entreprises, afin de renforcer leur valeur et de bonifier leur notation auprès de la Banque de France. Le but est de leur permettre de dégager des marges de trésorerie et d'éviter une nouvelle dégradation de leurs fonds propres en aggravant leurs déficits. leurs déficits. Les actifs incorporels, par exemple les fonds de commerce et les marques, représentent une grande part de la valeur de certaines entreprises, en particulier dans l'hôtellerie-restauration.

Cet amendement vise donc à harmoniser la durée de la plus-value de l'évaluation avec la durée de l'amortissement de l'immeuble, de façon que l'opération soit véritablement sans frottement fiscal. Cette disposition serait d'une immense aide pour les entreprises qui sont aujourd'hui

Guillaume Gontard. L'accompagnement des entreprises en difficulté engagées dans des opérations de cession-bail est légitime dans la période, particulièrement pour les plus petites d'entre elles, qui souffrent des conséquences économiques de la crise sanitaire. sur ce point, la mesure proposée, à l'instar des autres mesures gouvernementales, ne fait aucune distinction entre les entreprises, ni par taille, ni par secteur, ni selon leur santé financière ou encore leur impact environnemental. Dès lors, elle est susceptible de créer des effets d'aubaine et de bénéficier à des groupes bien portants versant des dividendes et engagés, par exemple, dans des pratiques d'évitement fiscal. De plus, on peut douter de la pertinence de la multiplication des mesures réglementaires et de leur intérêt comparé par rapport à des aides plus directes et plus ciblées. L'article 6 manque l'occasion d'utiliser les mesures d'urgence pour engager la transition écologique et sociale de notre économie. Le dispositif prévu à l'article 6 constitue un bon outil de relance, notamment pour éviter un ressaut immédiat d'imposition,

part, la mesure à d'autres crédits-bailleurs que les sociétés de crédit-bail- particuliers, sociétés cotées ou non, fonds d'investissement, etc. -, et, d'autre part, le bénéfice de l'étalement dans le cadre d'une cession-bail aux sociétés foncières. L'objectif est double : premièrement, faire jouer la concurrence avec un panel plus large d'acquéreurs, pour fixer le prix de cession le plus attractif et faciliter ainsi le refinancement des entreprises affectées par la crise sanitaire ; deuxièmement, en faire profiter les sociétés foncières touchées de plein fouet par la crise sanitaire et économique. L'amendement

L'article 7 instaure une suppression progressive sur trois ans du coefficient de 1,25 appliqué au bénéfice des titulaires de revenus passibles de l'impôt sur le revenu, qui sont soumis à un régime réel d'imposition et qui ne sont pas adhérents d'un centre de gestion ou organisme mixte de gestion agréé. Or les organismes de gestion agréés sont aujourd'hui la garantie de la fiabilité comptable et, bien souvent, de la viabilité de nombreuses de nombreuses petites entreprises. Dans le contexte de crise que nous connaissons, il semble prématuré de modifier le régime en vigueur.

entraînerait deux conséquences : d'une part, la perte pour la puissance publique d'un outil de sincérité fiscale et de lutte contre la fraude, qui existe depuis plus de quarante-cinq ans ; d'autre part, la disparition des OGA et des emplois induits. induits. La fréquence des contrôles fiscaux par l'administration fiscale concernant les petites entreprises est relativement faible aujourd'hui. Or, chaque année, 100 % des adhérents des OGA font l'objet d'un contrôle de cohérence et de vraisemblance de leur résultat fiscal, soit plus de 1,2 million de contrôles par an. Par ailleurs, il s'agit d'un faux cadeau fiscal, officiellement présenté comme une mesure de soutien à la trésorerie des TPE. En effet, ces entreprises bénéficient aujourd'hui d'un certain nombre de services coûteux

et met donc fin à l'avantage fiscal dont bénéficient les entreprises qui y adhèrent, engagées dans une démarche de transparence. Présentée comme une mesure de relance des TPE, cette disposition

remis en cause sans raison objective. Je ne veux pas, pour ma part, y voir l'action d'un lobby qui souhaiterait voir disparaître ces structures ...

le rapporteur général indique que, en 2014, la Cour des comptes aurait estimé que la plus-value des organismes de gestion agréés était difficile à établir.

imposable en cas de non-recours à un organisme de gestion agréé ou à un professionnel du chiffre. En revanche, une entreprise pourra toujours bénéficier du crédit d'impôt à raison de la cotisation acquittée pour adhérer à un OGA.

à la sagesse du Sénat

2006, avec pour objectif de fiabiliser la base fiscale de l'impôt sur le revenu en incitant les entreprises qui y étaient assujetties à recourir aux services d'organismes de gestion agréés.

ans après leur création, la contribution des organismes à l'amélioration de la connaissance des revenus non salariaux est difficile à établir », car « la proportion de redressements à l'issue d'un contrôle fiscal est identique chez les adhérents et non-adhérents ». Plus graves encore,

les rectifications effectuées par les OGA n'ont abouti à fiabiliser la base fiscale qu'à hauteur de 0,2 %, soit seulement 85 millions d'euros sur une base totale de 47 milliards d'euros

modique, pour montrer qu'ils luttent contre la fraude. Le président du Comité de déontologie parlementaire a très clairement résumé ce qui saute aux yeux de tout le monde : il n'y a aucune raison objective

En agriculture, la forme sociétaire gagne de plus en plus de terrain ; il faut donc accompagner ce mouvement et ne pas l'entraver par ce qui est perçu comme des contraintes fiscales. Il s'agit de faire en sorte que la disparition de la société absorbée dans le cadre de la fusion ne soit plus considérée comme une cessation fiscale d'activité. Cela implique l'imposition de toutes les sommes non encore imposées. Les opérations de fusion doivent être sécurisées pour que le reprenant sous la forme sociétaire ne reparte pas de zéro sur l'exploitation, s'agissant en particulier des engagements fiscaux de la société à travers des dispositifs suivants : la déduction pour investissement, la déduction pour épargne de précaution et la déduction pour aléas. Il serait plus logique de considérer la fusion comme une continuation de la société absorbée au sein d'une autre structure, à savoir la société absorbante. absorbante. L'amendement déposé par mon collègue Henri Cabanel vise à élargir le bénéfice du régime de faveur propre aux fusions de sociétés civiles professionnelles à l'ensemble des sociétés à objet agricole soumises à l'impôt sur le revenu, telles que les

le revenu ou à l'impôt sur les sociétés résulte d'un choix personnel de l'exploitant agricole. L'impossibilité, pour un exploitant soumis à l'impôt sur le revenu, de bénéficier, en cas d'apport du régime spécial des fusions, fait partie des critères à prendre en compte avant de déterminer le statut juridique et fiscal. C'est la raison pour laquelle nous sommes systématiquement défavorables à cet amendement.

comme vous, que les recherches publique et privée doivent travailler ensemble, qu'il n'y a pas d'opposition entre recherche appliquée et recherche fondamentale et que la participation des chercheurs publics à l'innovation privée est une nécessité. Nous partageons totalement

Nous constatons que, depuis dix ans ou plus, l'effort des entreprises en matière de recherche et développement stagne au niveau extrêmement faible de 1,44 % du PIB. Cette stagnation est due à une baisse de l'effort de recherche dans des secteurs stratégiques et essentiels : l'automobile, l'aéronautique, la pharmaceutique,

Notre problème est là : il réside dans la structure économique du pays. Le CIR, avec ses 6,5 milliards d'euros- la plus grosse niche fiscale -, ne change rien à cette structure. Il est un puits

étude de mars 2019 : elle démontrait que le crédit d'impôt recherche est une dépense fiscale efficace. J'ajoute que le CIR est souvent très attendu par la recherche publique.

Il bénéficie du super taux de CIR que l'Assemblée nationale vient de supprimer. Ce contre-exemple montre bien que le CIR est une absurdité en matière de recherche.

des projets d'investissements étrangers pour la recherche et développement.

à Mme Jacky Deromedi. Le soutien aux entreprises à travers le crédit d'impôt durant cette période incertaine est essentiel. Il est important, sans aggraver la situation financière dans laquelle se trouve notre pays, que nous puissions garder nos acquis, le temps que notre industrie voie venir des jours meilleurs. C'est la raison pour laquelle le présent amendement vise à supprimer l'article 8, afin de maintenir les dispositions initiales de l'article 244 B du code général des impôts relatives au crédit d'impôt pour les dépenses de recherche effectuées par les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles, supprimées par le Gouvernement, à mettre une condition suspensive : la révision du taux de crédit d'impôt sera effectuée dans le cadre d'une prochaine loi de finances, dans un délai de trois ans. L'amendement que nous avons adopté en commission tend à proposer une solution équilibrée puisqu'il ménage une période de transition pour les organismes de recherche, tout en sécurisant le crédit d'impôt recherche. Par ailleurs,

Gontard. Je suis d'accord avec ce qui a été dit sur le CIR : il faut repenser le système de manière globale. Un budget de réponse à la crise doit aussi être un budget efficace. Le crédit d'impôt recherche a été épinglé de nombreuses fois pour les abus qu'il permet.

car ces dépenses pourraient être bien plus utiles ailleurs pour faire face à la crise. Nous proposons donc de diminuer le taux du crédit d'impôt des grandes entreprises, celles dont les dépenses de recherche sont supérieures à 100 millions d'euros,

an, le CIR ayant été étendu aux grands groupes. Ainsi, en 2015, 14 000 entreprises avaient bénéficié du CIR, parmi lesquelles 42, soit 0,3 % des entreprises bénéficiaires, représentaient à elles seules 31 % des créances. Un rapport du Sénat avait pourtant démontré que 80 % des créations d'emplois permises par la recherche se faisaient dans les entreprises de moins de 500 salariés. Le crédit d'impôt recherche est devenu aujourd'hui un outil d'optimisation fiscale pour les grandes entreprises, bien plus qu'un soutien à la recherche. notre amendement permettrait de considérablement réduire les dépenses du CIR, tout en n'ayant aucun effet sur l'écrasante majorité des entreprises qui en bénéficient.

soit l'occasion d'une actualisation et d'une mise en conformité avec des règles et des instructions transmises par la Commission européenne, dans une logique de sécurisation. Cette dernière nous a amenés à procéder à un certain nombre de modifications, que nous considérons comme légères.

l'an passé, je vous ai mis en garde ici même contre le caractère sans doute difficilement soutenable, du point de vue des critères de Bruxelles, des super taux.

c'est ! C'est consciemment que tous, ici, nous laissons faire. C'est donc consciemment que nous laissons la porte ouverte à la fraude fiscale,

de la suppression du doublement d'assiette du crédit d'impôt recherche en cas de sous-traitance publique pour les petites et moyennes entreprises, en rétablissant à 50 % le taux de prise en compte forfaitaire des dépenses de personnel, qui avait été diminué à 43 % en loi de finances pour 2020, pour des raisons d'ordre budgétaire. En bonne coordination avec l'amendement tendant à repousser à 2023 la suppression du doublement d'assiette pour sous-traitance publique, la modification prévue par le présent amendement n'entrerait en vigueur qu'en 2023.

Mizzon. Le présent amendement a pour objet de mieux adapter le traitement fiscal des avances remboursables à la trésorerie des entreprises innovantes, en évitant que la fiscalité reprenne d'un côté ce que l'État a consenti de l'autre. Le droit en vigueur exige que les avances remboursables soient déduites de l'assiette du CIR le jour de leur perception et que leur remboursement soit intégré à cette assiette. En conséquence, les avances remboursables viennent limiter l'avantage fiscal lors de leur perception, mais elles l'augmentent lors du remboursement. Autrement dit, dans la période où l'entreprise a le plus besoin de trésorerie, celle-ci est diminuée, alors que, dans la période où elle n'en a plus forcément besoin, elle est augmentée. Afin de rendre le traitement fiscal des avances remboursables plus compatible avec la réalité économique des entreprises innovantes, l'amendement vise à neutraliser les effets de l'avance remboursable sur le crédit d'impôt recherche : ni déduction de l'assiette le jour de perception ni réintégration le jour du remboursement. Il s'agit d'une mesure de trésorerie sans effet sur les finances de l'État. Cet amendement tend également à améliorer le traitement fiscal des avances remboursables qui viendraient à être transformées en subventions, c'est-à-dire dont le remboursement ne serait plus exigé : aujourd'hui, la perception de l'avance entraîne une déduction de l'assiette du CIR demain, c'est au jour où l'avance serait transformée en subvention qu'elle viendrait limiter l'avantage fiscal. Il s'agit aussi de mieux adapter le traitement fiscal au profil de trésorerie des entreprises innovantes, ce sans effet sur les finances de l'État. Enfin, afin de s'assurer que cette modification ne donne pas lieu à des abus, un état de suivi des subventions remboursables paraît nécessaire.

Il se traduira néanmoins assez vite par un prélèvement sur le budget de l'État, estimé à 75 millions d'euros.

cette dernière a souligné que, si les avances remboursables sont comptabilisées en tant que dettes par les entreprises, elles constituent par ailleurs une aide publique du point de vue de l'État. Les intégrer dans l'assiette du CIR revient donc à accorder « une aide sur une aide Troisièmement, quand le projet de recherche aboutit, l'entreprise restitue le montant de l'avance, qui est alors prise en compte dans le calcul du

En effet, le rétablissement du régime antérieur à la réforme du crédit d'impôt opéré par la loi de finances pour 2008 conduirait à ce double avantage. Depuis cette réforme, les avances remboursables reçues par les entreprises en raison des opérations ouvrant droit au doivent être déduites des bases de calcul du crédit de l'année au cours de laquelle elles sont versées. Pour assurer la neutralité de la mesure au regard de leur CIR, les entreprises ajoutent les montants remboursés aux bases de calcul du crédit d'impôt de l'année au cours de laquelle les remboursements sont effectués. La disposition que vous proposez entraînerait un cumul

vise à obliger toute entreprise qui ferme un ou plusieurs sites en France à rembourser le montant perçu sur deux exercices au titre du crédit d'impôt recherche, dans la limite de la moitié de ce montant. Depuis plusieurs années, les fermetures d'entreprises justifiées non par une faillite, mais par le transfert d'activités dans un autre pays, soit pour réduire les coûts de production, soit pour une raison de stratégie commerciale, soulèvent la question de la responsabilité fiscale et de la justice sociale pour les salariés, face à un dispositif qui permet aux entreprises de déduire de l'impôt sur les sociétés 30 % de leurs investissements en recherche et développement et qui, rappelons-le, a un coût élevé pour les finances publiques, évalué à 6,27 milliards d'euros en 2017. Si la stabilité de ce dispositif fiscal, créé en 1983 et sanctuarisé depuis 2008, est reconnue comme un outil d'attractivité, certaines entreprises qui quittent le territoire français remplissent difficilement leurs obligations issues de la loi du 29 mars 2014 visant à reconquérir l'économie réelle, dite « loi Florange comme Nestlé, dans les Alpes-Maritimes, lors de la fermeture du laboratoire de recherche en dermatologie Galderma. Le Gouvernement a répété à plusieurs reprises depuis 2017 qu'il était prêt à faire évoluer le crédit d'impôt recherche en France, afin de responsabiliser les acteurs économiques qui y font appel. Ainsi, l'obligation de rembourser le montant perçu sur deux exercices, dans la limite de la moitié de ce montant, est réaliste et envoie un signal fort aux acteurs économiques qui ne perçoivent, dans le CIR, qu'un levier fiscal sans contrepartie sociale. L'objectif n'est pas de restreindre un outil d'attractivité ni de créer une « contrepartie ». Il s'agit de répondre à une réalité rapportée par la Cour des comptes dans une publication de 2013, qui souligne qu'« entre 2007 et 2011, le nombre d'entreprises déclarant du CIR a doublé, passant de 9 800 à 17 900 entreprises » et que leur créance fiscale est passée de 1,8 milliard à 5,2 milliards d'euros, « soit un quasi-triplement. Plutôt que de créer des contrôles fiscaux, qui nécessitent une logistique humaine et plus de financements publics pour un contrôle en amont systématique, cet amendement tend à fixer un cadre d'utilisation large du crédit d'impôt recherche, sans toucher au bénéfice fiscal final des entreprises.

Je souscris à l'objectif de moraliser le comportement des entreprises et suis donc sensible à l'intention des auteurs des amendements, qui cherchent à lutter contre les effets d'aubaine induits par le crédit d'impôt recherche. J'ai néanmoins deux sujets de préoccupation. D'une part, le droit européen fait obstacle à des dispositifs nationaux qui réservent le bénéfice d'un avantage fiscal aux seules dépenses réalisées dans le pays concerné. D'autre part, les créances du crédit d'impôt recherche sont couvertes par le droit de propriété, qui est garanti constitutionnellement. Les délais et conditions de la reprise rétroactive

de nouveau que les créances du crédit d'impôt recherche sont couvertes par le droit de propriété, constitutionnellement garanti. Les délais et conditions de la reprise rétroactive des créances font l'objet d'un encadrement très strict.

une évaluation générale de la recherche. La tâche d'instruire scientifiquement les rescrits fiscaux demandés par les entreprises pour bénéficier du CIR était jusqu'à présent confiée à l'Agence nationale de la recherche

Si la demande de rescrit concerne uniquement le caractère scientifique et technique d'un projet de recherche, elle peut être adressée directement au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Je m'interroge sur les intentions de l'auteur de l'amendement. S'agit-il de confier à cette autorité l'évaluation de la pertinence des rescrits adressés par les entreprises ? Le cas échéant, si les dépenses ne sont pas éligibles au CIR, CIR, l'administration fiscale et le ministère de l'enseignement supérieur le font savoir. S'agit-il de lui confier le soin de traiter les demandes de rescrit et donc de se prononcer sur le caractère scientifique et technique des projets de recherche ? Si tel est le cas,

explication de vote. Monsieur le ministre, je ne comprends pas ! Nous avons voté hier une loi qui fait du Hcéres l'organe fondamental de l'évaluation de la recherche scientifique

Je comprends que cette disposition, instaurée en 2004, pose problème au regard de la réglementation européenne sur les aides d'État, mais sa suppression pure et simple risque de porter atteinte au développement des partenariats public-privé, qui constituent pourtant un sous-jacent important du projet de loi de programmation de la recherche. Cela étant dit, mon cher collègue,

Le signal adressé par le Gouvernement est donc très contradictoire : les dirigeants d'établissements publics de la recherche à caractère industriel et commercial, pour lesquels la recherche partenariale est centrale, ont exprimé de vives inquiétudes auprès de beaucoup d'entre nous. La suppression de cette modalité de doublement d'assiette du CIR ne représente qu'une part faible du coût total du crédit d'impôt recherche pour l'État, mais risque d'avoir un impact négatif majeur dans cet équilibre entre recherche publique et privée. Cet amendement vise à repousser l'échéance du 1 janvier 2022 au 1 janvier 2024 et de permettre à l'État et aux acteurs concernés de faire réaliser une nouvelle analyse objective des avantages et limites du doublement prévu dans le dispositif CIR, de documenter précisément les conséquences de cette suppression, d'approfondir l'analyse juridique de la robustesse du nouveau dispositif au regard du droit communautaire, d'engager une réflexion sur l'ensemble des acteurs concernés- privés et publics -dans la perspective de trouver des solutions. Mon cher collègue Pierre Ouzoulias, vous avez l'air de dire que cela ne sert à rien, mais vous savez très bien que le développement de la recherche partenariale passe aussi par le soutien de structures comme les instituts Carnot, que nous soutenons et vous et moi, et dont la démarche originale consiste à analyser les besoins d'innovation des entreprises, puis à trouver les équipes de recherche capables d'y répondre. À notre satisfaction, le rapport annexé du projet de loi de programmation avait fait mention de la volonté de renforcer les dispositifs Carnot en faisant passer son abondement annuel 62 millions d'euros à 150 millions d'euros dans les prochaines années. Cette labellisation récente de nouvelles structures nécessite en effet une augmentation de la dotation de l'État, au risque de devoir attribuer une part plus réduite à chacun des instituts, ce qui entraverait inévitablement leur développement.

juridiquement le crédit d'impôt recherche. Comme vous l'avez souligné, et c'est également le travail de Jean-François Rapin, les organismes auront deux ans pour anticiper

à la lutte contre le changement climatique. L'une de ces transitions se caractérise par le passage d'une société fondée principalement sur les consommations abondantes d'énergies fossiles à une société plus sobre en énergie et faiblement carbonée. La fiscalité constitue un instrument de mise en oeuvre de ces objectifs.

amendements visent à lier le bénéfice du crédit d'impôt recherche au respect par les entreprises d'obligations environnementales.

techniques. L'article 8 prévoit un abattement exceptionnel applicable aux plus-values immobilières dans le périmètre d'une opération de revitalisation du territoire (ORT) ou d'une grande opération d'urbanisme

également de soutenir la construction dans les territoires concernés. Je soutiendrai à la fois l'article et l'amendement du rapporteur général visant à la remise d'un rapport

qui nous a proposé un second bilan sur l'imposition sur le capital- suppression de l'ISF et mise en place d'un prélèvement forfaitaire unique.

Mais il y a des symboles, mes chers collègues. Les Françaises et les Français, dans leur histoire, se sont parfois attachés aux symboles, pour résister, se rebeller et, parfois, poser la question du changement.

la création d'emplois. Le patrimoine polluant- avions privés, voitures de luxe et yachts -a également disparu de la base taxable, alors que le défi écologique est au coeur des préoccupations du Gouvernement. C'est suffisamment incohérent pour être inacceptable. Le présent amendement vise donc à réintégrer ce type de biens mobiliers corporels dans la base taxable. À la différence d'autres biens meubles par nature, ceux-ci connaissent un régime particulier qui les apparente à des immeubles. En effet, ils sont soumis à immatriculation, à partir de laquelle une publicité peut s'organiser. Tout comme un bien immeuble, ils peuvent faire l'objet d'une hypothèque ou d'un droit de suite, être identifiés et attachés à un « port d'attache La réintégration de ces biens dans l'assiette taxable de l'IFI, en plus d'être cohérente, serait bienvenue, compte tenu notamment de l'échec cuisant de la surtaxation des yachts votée dans le même temps, en 2017. Alors qu'un rendement de 10 millions d'euros par an était attendu

n'ont aucun intérêt à installer des jeunes sur les exploitations, ce qui constitue un véritable problème. L'exonération partielle ne constitue plus un un attrait suffisant pour les propriétaires de biens ruraux, qui sont très lourdement imposés au travers de différentes fiscalités.

devrait permettre l'installation de jeunes agriculteurs sur des exploitations, qui, sinon, connaîtraient une désertification.

pour des raisons constitutionnelles, il n'est pas possible de réintégrer uniquement les biens meubles dans l'assiette de l'IFI actuel. Je demande également

porter de 75 % à 100 % le taux de l'exonération des actifs fonciers agricoles de l'IFI, sans aucune condition d'exploitation par le redevable, pose assurément un problème d'égalité de traitement par rapport à la détention d'autres actifs. Quel est l'avis

Contrairement à ce que M. le ministre vient de dire, le Gouvernement n'a pas toujours exclu de revenir sur la mesure prise au début du quinquennat, conformément aux engagements de campagne. Voilà très exactement deux ans, en pleine crise des gilets jaunes, porte-parole du Gouvernement a affirmé, sous la pression politique qui s'exprimait du fait des injustices, notamment de l'injustice fiscale : « nous n'excluons pas de modifier le système

En réalité, l'effet économique de la suppression de l'ISF, ou plutôt de sa transformation en IFI, n'a pas été prouvé. En revanche, son effet sur l'explosion des inégalités

à la crise politique lancinante que traverse notre pays depuis des mois.

Avez-vous conscience du risque socio-politique que nous prenons à ne pas vouloir travailler à la réduction de ces écarts de revenus, alors que la paupérisation augmente et qu'une majorité de Français

fois, personne ne peut dire qu'il n'y aura pas besoin de faire contribuer le patrimoine. Personne ! S'il faut attendre d'être mis sous pression